L'article 1, comme cela a déjà été souligné, vise à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de trois ans. Le transfert s'effectue après une habilitation du procureur général. Pour certains actes, le directeur de la police municipale pourra agir directement après autorisation préalable du procureur de la République. Les agents de police municipale seraient également autorisés à établir des procès-verbaux lorsque cela ne nécessite pas de leur part un acte d'enquête, et ce pour une liste de contraventions définies. Il apparaît que le texte ne prévoit aucun mécanisme de contrôle des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire. En conséquence, cet amendement tend à proposer un double mécanisme de contrôle de l'action des agents de police municipale : d'une part, un contrôle par l'inspection générale de l'administration, qui sera défini par décret pris en Conseil d'État selon des modalités assimilables à celles qui sont mises en place pour la police nationale et pour la gendarmerie nationale contrôle par la voie judiciaire, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale prévoyant que les actes des agents de police municipale agissant comme officier de police judiciaire soient placés sous contrôle du procureur de la République.

Les nouvelles missions dévolues à la police municipale posent directement la question du lien entre les policiers municipaux, dans leurs fonctions de police judiciaire, et les administrations judiciaires qui en assument le contrôle.

barreaux, instaurant un double mécanisme de contrôle des agents de police municipale, à la fois par l'inspection générale de l'administration, dont le contrôle sera défini par décret pris en Conseil d'État selon des modalités assimilables à celles qui sont mises en place pour la police nationale et la gendarmerie nationale, et par un contrôle judiciaire, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale prévoyant que les actes des agents de police municipale agissant comme officier de police judiciaire soient placés sous contrôle du procureur de la République. Ces garanties nous semblent indispensables pour placer l'action de ces policiers municipaux dans le cadre de la mission judiciaire constitutionnellement définie. ? Mme Benbassa et Mme Cukierman proposent d'indiquer que les actes réalisés dans le cadre de l'expérimentation sont dirigés par le procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et de la chambre d'instruction. Cette partie de leurs amendements est déjà satisfaite par la rédaction actuelle de l'article 1. Elles proposent également de renvoyer à un décret le soin de définir les modalités du contrôle de l'action des agents de police municipale

à des dépistages soit du taux d'alcoolémie soit de l'usage de stupéfiants d'un conducteur présumé en infraction au code de la route ou impliqué dans un accident mortel ou ayant

Il s'agit d'autoriser les directeurs et chefs de service de la police municipale dans dix départements et pour une durée de six mois à soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une infraction grave.

amendement ne précisent pas la finalité de ces contrôles- les agents de police municipale n'étant pas compétents pour constater les infractions en question -ni les modalités de choix des dix départements concernés. En outre, les policiers municipaux peuvent déjà procéder à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, sous l'ordre et la responsabilité d'un officier de police judiciaire. J'entends bien qu'il s'agit d'être beaucoup plus pragmatique et d'aller directement

Demain, les policiers municipaux pourront, à l'instar des membres de la police nationale et des gendarmes, avoir accès à différents fichiers, en particulier celui des immatriculations. Toutefois, dans ces milliers de communes qui n'ont pas de police municipale, les maires sont dépourvus

Borchio Fontimp. Les remontées de terrain démontrent que certaines interdictions imposées par le législateur aux policiers municipaux sont de nature à les ralentir dans leur travail.

des policiers municipaux à quatre fichiers prioritaires : le système d'immatriculation des véhicules (SIV), le système national du permis de conduite (SNPC), le fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) et le fichier des personnes recherchées

Si cette proposition de loi prévoit d'accroître les missions de la police municipale avec l'objectif d'en faire l'une des composantes essentielles de la sécurité intérieure du pays, il est primordial de donner aux agents les moyens nécessaires pour répondre à l'exercice de leurs nouvelles compétences.

police municipale au fichier des objets et des véhicules signalés, ainsi qu'au fichier des personnes recherchées, lequel regroupe notamment les personnes interdites de manifestation, interdites de séjour et de territoire français, interdites de quitter le territoire français, interdites de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et les personnes faisant l'objet d'interdictions relatives à une peine alternative alternative à la prison. L'évolution, l'adaptation des polices municipales est primordiale pour endiguer l'insécurité grandissante dans les grandes agglomérations, notamment lors des manifestations, autorisées ou pas, où l'on retrouve encore et toujours les membres des Black Blocs ou autres milices d'extrême gauche, groupes organisés ultraviolents, bien connus des services de police et de justice et qui constituent une sorte de de génération sans identité, si ce n'est celle de détester tout ce qui est enraciné et qui porte un uniforme de police, qu'il soit national ou municipal. Ces associations, elles, ne sont pas dissoutes- allez savoir pourquoi ! La délinquance, les cambriolages et les agressions n'épargnent pas non plus les communes rurales. L'accès des policiers municipaux aux fichiers doit être pris en compte pour endiguer un ensauvagement qui frappe désormais la société tout entière. Puisque l'État semble vouloir se décharger d'une partie de sa fonction régalienne sur les communes, il doit aussi faire confiance aux élus locaux en leur accordant les moyens nécessaires- quand cela ne coûte rien. Ceux qui enfreignent la loi profitent trop souvent des trous béants dans le filet sécuritaire pour agir en toute impunité. La numérisation est un progrès, à condition qu'elle soit utilisée par toutes les forces qui peuvent permettre de rétablir l'ordre. L'utilisation de fichiers complets et rapides d'accès par la police municipale permettra un maillage territorial plus serré et donc plus efficace. La troisième force de sécurité du pays ne doit pas être la cinquième roue du carrosse, mais un véritable acteur du continuum de sécurité. En témoignage de soutien à nos polices municipales, désireuses de nouveaux moyens d'action pour assurer la sécurité, je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.

recommandation de la Cour des comptes. Ce serait un premier pas fortement apprécié de nos policiers municipaux. Parce qu'elle est un maillon essentiel dans la lutte contre toutes les formes d'insécurité, la police municipale doit aujourd'hui gagner en autonomie.

cette fois, à permettre aux policiers municipaux d'accéder à différents fichiers, notamment à celui des objets et véhicules signalés pour une durée expérimentale de cinq ans. Calquée sur la temporalité choisie par la commission des lois, cette expérimentation revêt un caractère nécessaire et est très attendue sur le terrain.

Ainsi, lors du contrôle d'un véhicule sur leur initiative, ils peuvent interroger les services de la police nationale pour déterminer si ce véhicule fait l'objet d'une inscription au fichier des objets et véhicules signalés. l'article 5 du décret sur le fichier des personnes recherchées leur permet d'être informés oralement d'informations qui y figurent, notamment afin de parer à un danger pour la population. Je rappelle également que notre ancien collègue

initiées par les polices municipales dans le cadre des statistiques nationales de la délinquance produites par le ministère de l'intérieur, afin de positionner la police municipale dans le paysage de la sécurité. Merci des indicateurs qui permettraient de mesurer l'activité des polices municipales et de mettre en place, en quelque sorte, des statistiques relatives aux saisines judiciaires initiées par lesdites polices. le rappelle, les polices municipales sont plurielles. Leur doctrine d'emploi dépend beaucoup de la volonté politique du maire, ainsi que de la nature de la délinquance sur le territoire. Il ne me semble donc pas très pertinent, au nom de l'autonomie des collectivités locales, d'introduire une mesure de leur activité,

Nous voterons bien évidemment cet amendement.

Mme Nathalie Delattre. L'un des objectifs de ce texte est de rapprocher la police municipale de la police et de la gendarmerie nationale, tant du point de vue de leurs fonctions que de leur capacité d'intervention.

d'entrer dans le corps de la police municipale, où ils sont, d'une certaine façon, rétrogradés de la fonction d'APJ adjoint. Cet amendement vise donc à redonner aux anciens gendarmes et policiers nationaux recrutés comme policiers municipaux les pouvoirs de police judiciaire pour lesquels ils ont reçu une formation

? Je me suis déjà exprimé sur ce point. Mme Nathalie Delattre propose d'attribuer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de police municipale qui étaient précédemment OPJ. Or le Conseil constitutionnel a déjà censuré l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire à des agents de police municipale. Si nous adoptions cet amendement, nul doute qu'il le censurerait à nouveau. Je ne peux donc pas y être favorable.

: La parole est à M. Stéphane Ravier. Cet amendement est une proposition de bon sens. Oui, cela arrive ! La commune est une réalité territoriale intrinsèque, mais certaines réalités, comme l'insécurité, ne tiennent aucun compte de ces limites administratives. Dans le cas d'une poursuite par un policier municipal d'un délinquant dangereux, c'est-à-dire d'un individu susceptible d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, puisque la prise en charge - et non plus en chasse - n'est plus autorisée pour pour tout autre acte de délinquance, l'adoption de cet amendement permettrait que l'interpellation puisse se faire sur le territoire d'une commune voisine par un policier municipal, dans le même cadre que lorsqu'il exerce ses fonctions dans les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. Les délinquants et les personnes en fuite font encourir un risque à toute la population et n'ont aucune frontière pour se déplacer et commettre leur délit. C'est pourquoi il paraît juste de ne pas contraindre les policiers municipaux de respecter un périmètre dont se moque bien la réalité. Si les délinquants ont une nationalité - certains en ont même plusieurs -, la violence n'a pas de passeport communal. Il est tout de même extravagant que les seules frontières infranchissables soient les frontières communales et que les seuls qui ne puissent les franchir soient les représentants des forces de l'ordre.

commission ? M. Ravier propose qu'on puisse autoriser un policier municipal à sortir de sa commune pour interpeller l'auteur d'un crime ou d'un délit. D'une part, je le rappelle, les policiers municipaux ne sont pas compétents pour interpeller les auteurs de crime ou de délit. Ils doivent en référer immédiatement aux officiers de police judiciaire compétents territorialement. D'autre part, vous l'imaginez aisément, si on laissait un policier municipal sortir de sa commune pour interpeller

à sa disposition un premier niveau de réponse pénale, qui prend la forme soit d'une indemnisation financière de la commune, soit d'une activité non rémunérée au profit de la commune. Seulement, la transaction proposée par le maire a jusqu'à présent rencontré peu d'écho dans les communes. En effet, ce dispositif peut sembler complexe à mettre en oeuvre, notamment pour des raisons juridiques. Dans les faits, la transaction est rarement mise en application. Aussi, par cet amendement, il s'agit d'assouplir et d'accélérer administrativement cette procédure. Pour y parvenir, il convient de repenser le rôle du procureur de la République dans le cadre de la procédure de transaction. Il ne serait plus nécessaire pour lui de l'homologuer. Le document lui serait simplement transmis. Il aurait toutefois la possibilité de s'y opposer dans un délai strict de quarante-huit heures et par une décision motivée. Une telle réforme serait également l'occasion de renforcer la confiance accordée aux maires et à leur rôle dans la répression de la délinquance. Quel ? L'intention de Mme Delattre est tout à fait louable puisqu'elle suggère que la transaction qui est proposée par le maire ne soit plus homologuée par le procureur, mais fasse l'objet d'une éventuelle décision. Je

Borchio Fontimp. Cet amendement tend à autoriser les agents de police municipale à réaliser des contrôles d'identité afin d'améliorer la sécurité de nos concitoyens et de renforcer leur confiance en l'État. un rapport de la commission des lois du Sénat sur les polices municipales indiquait déjà « que cette limite aux attributions des agents de police municipale peut susciter des difficultés dans la mise en oeuvre de leurs missions ». Constatant chaque jour l'implication de l'échelon local dans la sécurité du quotidien, j'estime qu'il serait opportun de faire évoluer la loi sur le sujet.

la commission des lois a opportunément modifié l'article 1 pour concilier l'exigence de bonne information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune avec la charge incombant au parquet. L'Assemblée nationale avait prévu une information systématique des maires pour les suites données aux infractions causant un trouble à l'ordre public et constatées par les agents de police municipale ou signalées au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Si cette idée peut paraître séduisante, elle n'est pas réaliste et serait sans doute contreproductive. En effet, comme j'ai pu le constater au travers des travaux que nous avons conduits avec Corinne Féret dans le cadre de notre rapport, l'information systématique des maires entraînerait une charge de travail démesurée pour les parquets. Je salue le travail de la commission des lois, qui a su trouver une position d'équilibre : il est légitime que le maire soit informé des suites judiciaires données aux infractions qu'il signale, dès lors qu'il en fait la demande au cas par cas et que cette information lui est nécessaire dans le cadre de ses fonctions. fonctions. Le garde des sceaux, que nous avons rencontré, a d'ailleurs appelé les procureurs à renforcer les relations institutionnelles avec les élus locaux dans une récente circulaire du 15 décembre 2020. Dans le cadre de nos travaux, nous avons reçu les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République, mais également le procureur de Valenciennes, lequel est parvenu à fluidifier les relations avec les quatre-vingt-deux maires de son ressort au travers notamment d'actions de formation dédiées aux élus locaux, la création d'une boîte aux lettres électronique gérée par ses soins et la mise en place de groupes de travail pour traiter des incidents qui perturbent la vie quotidienne des maires. Les parquets doivent répondre aux demandes du maire, et la relation maire-parquet doit être plus fluide. Le sentiment d'impunité doit être réduit au maximum, et les dépôts de plainte, traités dans les meilleurs délais. Ainsi, la réussite des politiques de sécurité sur le terrain permettra une articulation renforcée entre les élus locaux et le maillon judiciaire.

actuel issu de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique qui renforce déjà l'information du maire de manière équilibrée.

et municipales, qui éprouvent quelquefois le sentiment de travailler pour rien. Quel ? Tous ceux qui ont été maires savent bien que la procédure qui est prévue dans les textes n'est pas systématique.

cela était précisé dans ce texte, le continuum de sécurité suppose aussi que le maire soit informé quand il l'estime nécessaire des suites d'une affaire. L'articulation entre le procureur et le maire

faits, peu respectées. Par ailleurs, nombre de ces infractions font l'objet d'un classement sans suite sans qu'il soit indiqué aux maires les motifs ayant conduit à cette décision.

Il conviendrait donc que le maire soit informé systématiquement des raisons pour lesquelles une infraction, qu'il l'ait ou non signalée, a été classée sans suite. Le présent amendement vise ainsi à étendre l'obligation d'indiquer au maire, lorsque celui-ci interroge le procureur de la République, les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient un classement sans suite, que l'infraction soit constatée par la police municipale, par la police nationale ou par la gendarmerie. Quel

prévoit que le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune, tant par les agents de la police municipale que par les forces de police nationale et de gendarmerie.

tout au long de l'exécution de leurs missions. En effet, l'extension de leurs prérogatives justifie à nos yeux un encadrement et des garanties supplémentaires. Nous demandons donc,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 2 apporte une modification subtile, mais aux conséquences non négligeables au code de la sécurité intérieure.

Nous doutons de l'utilité d'une telle disposition, et une fois de plus, nous nous opposons à ce glissement sécuritaire. Si la volonté de ce gouvernement est d'étendre les champs d'intervention de la police municipale, cela doit être fait dans le sens de l'accompagnement, du dialogue, de la médiation et de la participation citoyenne à la paix collective et à l'apaisement des conflits, et non pour créer encore plus de contrôle et de surveillance des citoyens.

que les polices municipales procèdent à des inspections visuelles de bagages et à des palpations lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, et qu'elles accèdent ainsi à des prérogatives propres à la police nationale. À l'époque, nous nous étions opposés à cette notamment parce que c'est un cadeau empoisonné pour les communes qui dépensent de plus en plus pour assurer la sécurité de manifestations sur leur territoire. Cet article

: il n'y a plus de manifestations sportives ou presque, plus de manifestations culturelles- ce qui suscite d'ailleurs beaucoup de mouvements de contestation en ce moment -, plus de manifestations associatives.

s'agit d'un amendement de suppression. L'article 2 de la proposition de loi permet aux agents de police municipale affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité, quelle que soit la taille de la manifestation, alors que ce n'est possible dans le droit actuel que pour les manifestations d'au moins 300 spectateurs. Ce seuil, jugé très restrictif par les auteurs de la proposition de loi, est supprimé. D'apparence anodine, la suppression du seuil de 300 spectateurs n'en soulève pas moins une difficulté en ce qu'elle méconnaît le respect des principes de finalité et de proportionnalité. Les opérations de vérification- palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages -auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises pour accéder ou circuler dans le périmètre de la manifestation sont justifiées par des raisons de sécurité liées à l'importance du nombre de personnes qu'elles sont susceptibles d'attirer. La finalité de la mesure est circonscrite et ne peut s'appliquer à n'importe quel rassemblement de personnes dans le cadre d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle, car entrent en ligne de compte le droit d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée. C'est dans le même esprit que ce critère s'impose pour conditionner la mise en oeuvre des périmètres de protection. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, un périmètre de protection ne peut en effet porter que sur un lieu ou un événement exposé « à un risque d'actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation En outre, l'article 2 est une source d'insécurité juridique, alors que la finalité recherchée et les catégories d'agents habilités à procéder aux vérifications sont identiques. Cette mesure reviendrait à dissocier les manifestations rassemblant un grand nombre de personnes de celles qui sont mineures, selon qu'elles se déploient dans le cadre d'une manifestation ou dans le cadre d'un périmètre de sécurité.

Tous les collègues élus locaux savent bien que tout dépend de la nature des manifestations, du contexte dans lequel elles se déroulent, du type de personnes qui peuvent les fréquenter, etc. C'est pourquoi nos collègues députés ont voulu supprimer ce seuil à juste titre.

et manifeste, l'IPM. Dès son origine, le dispositif de lutte contre l'ivresse publique a été conçu comme comportant une mesure de police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger les personnes. Actuellement, le placement en chambre de sûreté ne peut être décidé que par des agents relevant de la police ou de la gendarmerie nationale. À ce titre, le transport à l'hôpital de la personne recueillie en état d'ébriété sur la voie publique

justifiera, à terme, un transfert complet de compétences des policiers nationaux et de gendarmerie aux policiers municipaux qui ne disposent ni des moyens ni de la formation adéquate. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression du présent article.

poursuivrai donc l'exposé des difficultés que peut poser l'article 3. La procédure d'interpellation pour ivresse publique manifeste fait l'objet de nombreux débats, notamment d'un rapport très fouillé de quatre inspections générales- des affaires sociales, de l'administration et des services judiciaires -qui pointe certains dysfonctionnements. Cet excellent rapport, dont je vous recommande la lecture ou la relecture, monsieur le ministre, fait état d'une très grande hétérogénéité dans la mise en oeuvre de la procédure la présentation de l'interpellé au corps médical n'est pas systématique ; les actes de procédure et la réponse judiciaire ne sont pas homogènes ; la formation des personnels est limitée. La conclusion de ce rapport est assez limpide : « Il Il n'a pas paru [ ...] conforme à la logique française de répartition nationale des pouvoirs, de confier à des polices municipales le pouvoir régalien de retenir une personne contre son gré, l'État étant le meilleur garant de la neutralité et de l'impartialité des interventions publiques. » On ne peut pas être plus clair. Nous sommes dans le coeur du présent débat : le désengagement de l'État et le transfert de nombreuses compétences de police judiciaire aux polices municipales entraîneront à n'en point douter des disparités dans l'application de leurs prérogatives et,, des inégalités de traitement sur le territoire national. Interpeller une personne en état d'ivresse peut avoir des conséquences imprévisibles et potentiellement dangereuses : les bons gestes, la modération, la désescalade sont indispensables pour circonscrire le risque à un minimum.

Pourtant, la création d'une police municipale à Paris est indispensable et urgente. Elle est indispensable pour permettre à la préfecture de police de recentrer ses missions sur le maintien de l'ordre, la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Elle est urgente parce qu'il faut répondre à l'insécurité des Parisiens,

de ne pas inclure dans la formation initiale des policiers qui exercent à Paris un apprentissage au tir, dans le but de professionnaliser encore davantage ces agents. En France, plus de la moitié des policiers municipaux sont désormais munis d'une arme à feu. Les forces de police municipale doivent avoir les moyens de se défendre et de défendre leurs concitoyens face aux multiples dangers auxquels ils sont confrontés. Il serait irresponsable de leur refuser cette protection.

opéré, l'an dernier, un revirement visiblement stratégique pour tenter de masquer un très mauvais bilan en matière de sécurité à Paris. La priorité est désormais de créer une police municipale de plein exercice en mettant fin, autant que faire se peut, à l'exception parisienne en matière de répartition des pouvoirs de police. Nous espérons qu'à l'instar de nombreuses polices municipales, les agents parisiens pourront disposer d'un équipement adéquat, constitué de gilets pare-balles, de caméras-piétons, de radios localisées, d'une flotte de véhicules sérigraphiés, équipés

un handicap considérable pour assurer les missions de sécurisation et de tranquillité publique que réclament pourtant de nombreux Parisiens. En effet, Paris n'est pas un espace comme les autres. Capitale politique, institutionnelle et culturelle, la ville est aussi le lieu de résidence de plus de 2,2 millions d'habitants, le lieu de transit quotidien de millions de Franciliens et aussi celui de séjour de dizaines de millions de touristes.

qui entretient une confusion préjudiciable entre les missions de police municipale et les missions de sécurité publique de la police nationale.

à entretenir ce désengagement. Les propos que j'entends sur les missions qui devraient être celles de la police municipale parisienne, et sur la possibilité de son armement, contrairement

Nous sommes globalement d'accord avec l'idée d'un conseil de concertation entre les élus parisiens et le préfet de police.

les maires de chaque arrondissement ou leurs représentants, et le préfet de police de Paris. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d'emploi de la police municipale.